Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre aux voix successivement. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application de l'accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu,

pour procéder à une audience à distance et derrière un écran. Nous l'avons déjà exprimé maintes fois : nous sommes contre cette justice dématérialisée, qui finira, pour des motifs économiques évidents, par s'étendre à toutes sortes d'audiences. En l'espèce, son usage est d'autant plus contestable qu'il s'applique aux détenus provisoires. En effet, la détention provisoire est déjà largement dérogatoire au droit commun et plus que discutable, dans la mesure où, pour faire simple, des personnes non jugées sont mises derrière les barreaux.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux,

pas d'ordonnance motivée, pas de débat contradictoire ! Certes, on a évoqué le fait qu'il suffirait, dans ce cas, à la personne concernée de demander la mainlevée de la mesure, mais c'est autre chose.

une vigilance sur les conditions de restriction de la liberté d'aller et venir des personnes doit s'imposer. C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.

s'agissant d'une mesure de contrainte qui est moins attentatoire à ces droits que le placement en détention provisoire. La possibilité d'agir et de contester la mesure à n'importe quel moment constitue de ce point de vue une forme de protection. La commission émet

de la justice. Le manque de lisibilité des règles applicables à l'assignation à résidence sous surveillance électronique lors de la clôture de l'instruction avait notamment été avancé

absolument pas sur la nécessité de prolonger l'assignation à résidence tous les six mois au cours de l'instruction ; elle prévoit uniquement que cette prolongation n'est pas nécessaire après la clôture de l'instruction et le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction de jugement. En outre,

tombe à merveille, puisqu'elle me permet de préciser que le budget que nous proposons pour le ministère de la justice nous permettra de recruter 1 500 conseillers d'insertion et de probation supplémentaires.

Mme la garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir l'extension du recours à la visioconférence en matière de prolongation de la détention provisoire. projet de loi, tel que je l'ai déposé, prévoyait de supprimer la nécessité de l'accord de la personne détenue pour l'utilisation de la visioconférence lors des débats en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention. commission des lois a supprimé ces dispositions. Le Gouvernement estime cependant qu'il est indispensable de favoriser, dans certains cas, le recours à la visioconférence. Nous avions évoqué ce sujet lors de la discussion générale ; vous vous en souvenez sans doute, Il apparaît en effet nécessaire de remédier aux importantes difficultés que rencontrent les juridictions et qui sont liées à l'impossibilité d'assurer l'extraction de la personne détenue et donc sa présentation devant le juge dans les délais impératifs de comparution prévus par la loi, ce qui entraîne parfois des remises en liberté qui semblent injustifiées. En 2017, plus de 12 000 extractions judiciaires n'ont ainsi pas pu être prises en charge par l'administration pénitentiaire, soit près de 15 % des réquisitions d'extraction judiciaire. Le Gouvernement a toutefois pris en compte- je tiens à le souligner -les observations faites par les représentants nationaux de la profession d'avocat, notamment le Conseil national des barreaux, ainsi que par le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats, organisations qu'il a entendues dans le cadre de la concertation conduite après le dépôt du projet de loi. Je reconnais ainsi que la visioconférence ne doit pas pouvoir être utilisée sans l'accord de la personne détenue pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire. C'est uniquement pour les débats qui concernent la prolongation de cette détention que l'exigence d'un accord de la personne devrait être écartée. Nous avons donc fait évoluer notre texte. Tel est l'objet du présent amendement, qui tend l'accord de la personne pour les débats sur le placement en détention, mais l'exclut en revanche pour sa prolongation. Il me semble qu'il s'agit d'une solution raisonnable et équilibrée.

il me semble assez raisonnable d'essayer de préserver du temps pour les forces de sécurité. Quant à la question purement juridique, ou de préservation des libertés, et dans le prolongement de l'intervention de M. le rapporteur,

place le système de visioconférence uniquement pour le renouvellement de la détention provisoire, et non pour le premier placement.

communiquez par visioconférence, cela pose problème ! Or nous sommes en train d'améliorer considérablement le parc de la visioconférence, de sorte qu'il n'y ait plus de difficultés. C'est un point important. Quatrièmement, ce système fonctionne déjà.

sur d'autres personnes mêlées à l'affaire, auquel cas la bonne tenue de l'enquête justifie cette détention provisoire. Je crois profondément que la distinction que vous faites entre la première mise en détention

on peut avoir une appréciation qui justifierait que la procédure soit relativement plus souple que pour la prolongation. la prolongation. Celle-ci, en quelque sorte, est plus grave que la mise en détention. En effet, quand vous avez été deux mois en détention provisoire et qu'on renouvelle celle-ci pour plusieurs mois supplémentaires, cette détention prend une autre tournure c'est presque une peine qui s'applique sans le nom. Je ne vois donc pas pourquoi la procédure devrait être plus souple pour le renouvellement que pour la première mise en détention provisoire. Je dirais même que, si l'on devait distinguer entre les deux décisions, il faudrait que la procédure soit plus souple

La difficulté qui demeure, madame la ministre, c'est le risque de facilité. Lorsque la personne ne sera pas devant le juge et que l'enquête sera toujours en cours,

Dans sa rédaction actuelle, l'article 122-1 du code pénal établit en effet une distinction théorique entre l'abolition du discernement et du contrôle des actes d'une personne et l'atténuation du discernement ou entrave au contrôle de ses actes. Dans le premier cas, cela se traduit par la reconnaissance d'une irresponsabilité pénale, mais dans le second cas la responsabilité pénale peut être engagée, avec une adaptation des peines prononcées le cas échéant. Si cette distinction est satisfaisante sur le plan théorique, dans la pratique il apparaît qu'elle reste difficile à établir par les neuroscientifiques et les psychiatres, en particulier concernant les états de crise des personnes malades psychiques. Il existe un consensus pour préciser que, dans ces cas- crise d'hallucinations, violentes angoisses, sentiment de persécution, etc. -, la capacité d'exercer sa pleine volonté dans le contrôle de ses actes est particulièrement affectée, en plus du discernement. Le présent amendement tend donc à préciser les circonstances dans lesquelles l'irresponsabilité pour trouble psychique ou neuropsychique peut-être constatée. De façon plus globale, une réflexion approfondie sur les failles du système actuel de prise en charge de ces personnes doit être conduite,

le fond, dans la situation actuelle, le trouble grave du discernement justifie une diminution de la peine, comme le Sénat l'a d'ailleurs réaffirmé en adoptant la loi Taubira de 2014, mais non une totale irresponsabilité pénale,

que les personnes atteintes de maladies psychiques n'ont pas leur place en prison. Selon l'Observatoire international des prisons, près de 17 000 détenus en France présentent des troubles et des maladies psychiatriques. C'est plus que le nombre de places que le Gouvernement s'était engagé à construire. En outre, en détention pénitentiaire, à l'exception des unités hospitalières spécialement aménagées, les

parmi les mesures alternatives à l'emprisonnement, le sursis probatoire incluant l'observance de soins psychiatriques adaptés. Cette mesure permettrait de favoriser l'insertion ou la réinsertion des personnes et de prévenir le risque de récidive.

et à ce que peuvent faire les personnels médicaux dans les prisons. En effet, si un détenu placé en hôpital psychiatrique a l'obligation de suivre les thérapies qui lui sont proposées,

qui a été instaurée en 2004 afin de désengorger les tribunaux correctionnels. Cette procédure ne peut être mise en place que sous certaines conditions, notamment la reconnaissance des faits de la part de la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de « plaider-coupable » à la française.

par an au niveau national-, essentiellement car elle ne correspond pas à un besoin véritable, les informations judiciaires auxquelles elle est susceptible d'être appliquée étant de fait très rares. La CRPC, mode de jugement dégradé et superficiel, apparaît en effet peu compatible avec le niveau de gravité et de complexité que suppose par principe le recours à une information judiciaire. Le projet de loi prévoit néanmoins de renforcer ce mode de jugement en permettant au au parquet de se dispenser du travail de règlement de la procédure et au juge d'instruction d'éviter la rédaction d'une ordonnance de renvoi motivée- une exigence pouvant pourtant considérée

l'utilité et qui est de nature à créer de lourdes difficultés dans les quelques dossiers pour lesquels elle serait utilisée, dans l'espoir de gains de temps

En particulier, l'amélioration du mécanisme du règlement contradictoire, qui s'appliquera si une partie l'a demandé et non de manière systématique, a vocation à être maintenu, afin de raccourcir les délais de l'instruction dans un souci d'efficacité et de bonne administration de la justice- nous évitons d'ailleurs la systématisation du délai de trois mois en prévoyant un délai de quinze jours. De même, l'uniformisation du délai d'appel du procureur de la République des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction sur ceux du procureur général et des autres parties nous semble pleinement justifiée. Enfin, nous proposons de mettre en place une passerelle

il n'en demeure pas moins que le respect du contradictoire constitue une pièce maîtresse dans le déroulement du procès pénal, car il est la condition de l'exercice effectif des droits de la défense. Dans le droit en vigueur, le juge d'instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République et en aviser en même temps les parties et leurs avocats aussitôt que l'information lui paraît terminée. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ce règlement définitif est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, pour formuler des demandes ou pour présenter des requêtes. À l'expiration de ce délai, les parties ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. L'article 36 du texte initial du présent projet de loi donne un délai de dix jours aux parties pour annoncer si elles souhaitent recourir aux mécanismes de règlement contradictoire de l'instruction ou y renoncer. On escompte que les parties ne recourent à ce mécanisme que si elles estiment qu'il présente un intérêt. Mais, en pratique, le mécanisme du règlement contradictoire ne s'appliquera que si une partie l'a demandé et non de manière systématique. Outre que le dispositif retenu par l'article 36 complexifie la procédure, ce qui nous semble contraire à l'objectif du projet de loi, le mécanisme envisagé oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire, donc à la protection du justiciable. La commission des lois a porté ce délai de dix à quinze jours. Nous estimons qu'il serait plus raisonnable de laisser aux parties un délai de quarante-cinq jours, afin que celles-ci disposent de plus de temps pour prendre position.

Il me semble que porter ce délai à quarante-cinq jours serait complètement excessif. En effet, il excéderait ainsi le délai d'un mois qui est accordé aux parties pour présenter leurs réquisitions, observations et demandes dans le cadre du dossier qui concerne une personne détenue.

délais de règlement, car, dans la plupart des dossiers, il n'y a pas de demande d'actes. Le délai de trois mois allongeant inutilement la procédure, nous souhaitons vraiment en rester au délai de quinze jours qui est proposé.

afin d'étendre la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant à juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d'identité, tout en lui permettant de statuer à juge unique, le cas échéant sans audience, pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s'imposer. Ces dispositions constituent selon nous des simplifications cohérentes. la rigidité des règles d'examen en formation collégiale des requêtes en annulation ne se justifie pas lorsque la nullité est évidente. Ces simplifications sont d'ailleurs très attendues par les acteurs du droit, compte tenu de la longueur des délais de traitement par la chambre d'instruction, du fait de son encombrement. Cependant, pour tenir compte des inquiétudes de la commission des lois, il est proposé que, si l'auteur de la requête le demande, celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

la procédure dite « du plaider-coupable », le projet de loi prévoyait que, lorsque la proposition émanait du procureur de la République, les parties disposaient d'un délai de dix jours pour se prononcer. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables. Cette solution permet au parquet de se dispenser du travail de règlement de la procédure et au juge d'instruction d'éviter la rédaction d'une ordonnance de renvoi motivé. Or le règlement nous semble constituer un indispensable travail de synthèse et d'analyse de la procédure. Nous avions déposé en commission un amendement de suppression de cette mesure, qui a été adopté par la commission des lois.

L'article 36 du projet de loi allège la charge de la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale. Il étend dans trois matières la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant à juge unique,

Présenté il y a quelques mois par le Gouvernement comme un premier pas vers la décriminalisation de l'usage des stupéfiants, qui viendrait remplacer les peines de prison

le bon sens devrait primer. Plutôt que la répression, une véritable politique de santé publique et de prévention devrait être mise en place. Plutôt que d'enfermer les consommateurs victimes d'addiction, accompagnons-les Depuis plusieurs années maintenant, je milite pour la légalisation contrôlée du cannabis- j'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens -, ainsi que la décriminalisation des autres drogues comme l'héroïne, la cocaïne ou le crack. Nous ne saurions mettre tous les stupéfiants sur le même plan, comme le fait notre droit. Le cannabis a déjà fait l'objet d'une légalisation contrôlée dans certains pays européens et États fédérés américains, ainsi qu'au Canada, pour la consommation récréative aussi bien Malgré la répression accrue de la consommation du cannabis dans notre pays, le nombre d'utilisateurs augmente vertigineusement d'année en année. On aurait pu au moins espérer la dépénalisation du cannabis, qui est déjà effective dans la grande majorité des pays européens. l'amende délictuelle ne constitue nullement une dépénalisation, bien au contraire. Quant aux autres stupéfiants, ils créent dans tous les cas une dépendance et nuisent fortement à la santé de leurs consommateurs. Il est urgent d'accompagner ceux-ci, et de la meilleure manière. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait donné quelques gages en faveur de la légalisation du cannabis. Aujourd'hui, il rétropédale et traite la question aux antipodes de ses promesses antérieures. envisager de meilleur moyen de contrôler une consommation que de la rendre légale afin de la réguler et d'en prévenir les risques tout en s'adonnant à la prévention en général et à l'accompagnement des addicts C'est pourquoi nous enjoignons l'exécutif à mener une réflexion en la matière. Il est temps de poser avec courage et pragmatisme la question de la légalisation contrôlée du cannabis. La parole Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, sous le titre « Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire », l'article 37 crée trois groupes d'amendes forfaitaires délictuelles, qui s'ajouteraient aux deux cas déjà prévus par la loi de 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI siècle. L'amende forfaitaire délictuelle constitue à mon sens une une négation absolue du principe d'individualisation de la peine, en ce qu'elle réduit l'acte de juger à l'application de tarifs à la seule appréciation des forces de l'ordre, sans intervention préalable de magistrats. Selon le Syndicat de la magistrature, c'est d'autant plus grave que l'on nous propose ni plus ni moins d'étendre ce dispositif d'amende forfaitaire à trois nouvelles infractions, dont la principale est l'usage de stupéfiants, alors même qu'il reste purement et simplement inapplicable en pratique, faute de mesures réglementaires d'application, en raison d'obstacles juridiques et techniques non résolus. De plus, loin de l'ambition de clarification affichée, ce projet de loi sème la confusion sur un certain nombre de points. Ainsi, il y a une réelle incohérence entre le montant des amendes forfaitaires prévu par le projet de loi et les peines délictuelles encourues. Par exemple, l'amende forfaitaire pour la conduite sans assurance- 500 euros -est plus lourde que celle qui est prévue pour la vente d'alcool à un mineur- 300 euros -, alors que c'est l'inverse concernant leurs peines délictuelles, respectivement 3 750 euros et 7 500 euros. De la même façon, l'article L. 3353-5 du code de la santé publique prévoit qu'aucune peine ne sera appliquée au prévenu qui peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade ». de l'application de cette disposition en cas de procédure de forfaitisation ? En outre, je tiens à le souligner, la mise en place d'une amende forfaitaire pour usage de stupéfiants n'empêcherait aucunement les poursuites directes devant le tribunal correctionnel et ne constituerait donc pas un allégement de la répression ni une simplification : elle serait plus vraisemblablement de nature à « élever significativement le niveau de répression de l'usage de stupéfiants Cela va clairement à l'encontre du rapport de la mission d'information parlementaire du mois de janvier 2018, qui recommande la contraventionnalisation de l'usage de stupéfiants au regard des moyens insuffisants accordés à la justice pour traiter ce délit. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement

un net recul quant à la santé, aux avancées des politiques de réduction des risques et aux droits des usagers et usagères de drogues, qui demeurent les oubliés des politiques publiques qui les concernent. En réalité, cette mesure d'extension de l'amende forfaitaire délictuelle au délit d'usage de stupéfiants n'a d'autre finalité que de poursuivre et d'affirmer la politique du chiffre et de faciliter la répression, en rendant la procédure plus expéditive, en faisant fi des pratiques diverses- pour la plupart non problématiques -, de la consommation de stupéfiants, et cela bien évidemment en en passant sous silence les enjeux sanitaires. Pourtant, un consensus se dégage, y compris en France, pour réduire la pression pénale. environnemental, publié au mois de juin 2015 pointe les limites de la politique répressive, souligne la nécessité de lever les stigmatisations qui pèsent sur les usagers et usagères de drogues et plaide en faveur de l'ouverture

place policiers et gendarmes dans la position d'évaluer la situation sociale et sanitaire d'une personne, dans un contexte qui ne permet pas de prendre en compte la complexité des parcours, des trajectoires et des risques associés à la consommation.

au contexte de la pratique, aux facteurs de vulnérabilité de la personne, à la fréquence et à la quantité, bien plus qu'au caractère licite ou illicite des substances. Mes chers collègues, sachez que, avec ce choix, la France ferait toujours partie des six pays européens continuant de sanctionner l'usage de cannabis par une peine de prison ferme,

Je sais qu'il est compliqué d'avoir une échelle de peines performante pour un usage qui est aujourd'hui devenu un effet de société, un fait de voire un snobisme entre copains, une façon de se prouver, lorsque l'on est adolescent, que l'on est un homme, fort, costaud, et que l'on peut ainsi entrer dans le monde des adultes.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, cet article traite de l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants. Cette mesure a été présentée par le ministre de l'intérieur comme une réponse permettant de simplifier le travail des forces de l'ordre et de la justice et visant à automatiser les peines en la matière. le principe d'individualisation de la peine est ici bafoué, et la mesure octroie un pouvoir arbitraire aux forces de l'ordre chargées d'appliquer la contravention. pourront de ce fait sanctionner sans limites, au plus grand mépris des droits des personnes suspectées. En plus d'augmenter les inégalités des citoyens devant la loi, une telle mesure est dénuée de toute réflexion sur les questions relatives à la santé publique, pour ce qui a trait à la prévention et au traitement de l'addiction. Le seul effet de l'amende sera d'aggraver par une sanction pécuniaire une situation souvent déjà précaire nous savons que les comportements de consommation sont diversifiés et divergent entre les milieux paupérisés et les milieux mondains. Ce dispositif, en plus d'accroître le millefeuille législatif en matière de répression de l'usage des stupéfiants, semble inefficace, compte tenu de l'impossibilité juridique d'appliquer une amende forfaitaire délictuelle pour les mineurs, qui, pour certains

Cette mesure, mes chers collègues, est quelque peu rétrograde. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'alinéa 2 de cet article.

Mme Brigitte Micouleau. Cet article prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants. Il s'agit du même principe que les amendes forfaitaires délictuelles pour la conduite sans permis ou sans assurance voté dans la loi de modernisation de la justice du XXI siècle. Or il est prévu ici d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire, y compris en cas de récidive. Cet amendement vise donc à supprimer la procédure de l'amende forfaitaire en cas de récidive, afin de ne pas affaiblir la fermeté de la réponse pénale et de ne pas donner un sentiment d'impunité. Quel

qui, aujourd'hui, fument dans les lieux publics. La forfaitisation est précisément destinée à cela : dans les rues, aux sorties des écoles, cette procédure d'amende forfaitaire délictuelle nous permettra de résoudre ce problème. cette amende forfaitaire donnera lieu à une instruction générale des procureurs locaux pour sanctionner efficacement les consommateurs qui, aujourd'hui, font l'objet de simples rappels à la loi. Par conséquent, nous aurons une gamme supplémentaire, qui sera sans doute beaucoup plus dissuasive. Je crois que c'est ce que nous avons

n'empêche en aucune manière les réponses pédagogiques et sanitaires pour les toxicomanes habituels ou pour des drogues un peu plus dures. La direction des affaires criminelles et des grâces, dont le directeur se trouve à mes côtés, rappellera en effet au parquet leur appartiendra de diffuser des instructions spécifiques, qui viendront encadrer la mise en oeuvre de cette procédure et qui leur permettront de contrôler ce type de profil, afin que, au lieu d'une amende forfaitaire, soit mise en place une réponse sanitaire, sociale, pédagogique correspondant à un certain type de consommateurs.

Cette diversité nous permettra d'individualiser les réponses face aux différents types d'infractions auxquelles nous aurons affaire.

Cet article maintient la pénalisation de l'usage de stupéfiants, mais ouvre la possibilité d'éteindre l'action publique, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Ces modifications ne marquent pas un changement fondamental d'approche, pourtant nécessaire, mais ouvrent des risques de discrimination sociale entre ceux qui auront les moyens de payer les amendes et les plus démunis, qui ne le pourront pas. De plus, le maintien au sein du code de procédure pénale d'un stage de sensibilisation donnerait la possibilité de responsabiliser et sensibiliser les consommateurs de produits stupéfiants aux risques sanitaires et sociaux, en leur proposant une réponse éducative, ou en plus, du paiement d'une amende minorée. La seule création de l'amende forfaitaire aboutit à un véritable permis de consommer sans amener à une réflexion en termes de santé publique, alors que le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants de l'usage de produits stupéfiants permet d'engager une réflexion sur les dangers de la consommation et crée des passerelles vers la démarche de soins.

Cet article prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs et usage de stupéfiants. Il s'agit là de l'une des propositions du rapport Beaume et Natali, qui évoque aussi les délits d'occupation des halls d'immeuble. Il est donc proposé de fixer le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'occupation des halls d'immeuble selon le barème suivant : 300 euros, minorés à 250 euros et majorés à 600 euros. à 600 euros. Quel est l'avis de la commission ? On comprend parfaitement le sens de cet amendement. En revanche, le véhicule juridique qui est proposé est moins bien adapté que l'ordonnance pénale.

que pour les délits dont la constatation relève d'une forme d'évidence. C'est par exemple le cas pour le délit de vente d'alcool aux mineurs, où, au fond, il suffit d'établir que l'acheteur est mineur et que le produit vendu est de l'alcool. Ce n'est pas le cas pour le délit d'occupation illicite d'un hall d'immeuble, qui nécessite que soit établi le trouble causé à autrui, et ce n'est possible qu'à la suite d'investigations complémentaires, telles que des auditions.

Il nous semble que la commission va trop vite en proposant une généralisation sans évaluation approfondie des cas dans lesquels pourrait se pratiquer l'amende

il serait permis de forfaitiser des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ou encore le délit de dégradations légères par inscriptions sur les façades, véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, ce qui ne semble pas

à opérer ; pour les autres infractions, c'est plus compliqué, parce qu'il faut recueillir des preuves et procéder à des constatations, ce qui n'est pas toujours adapté. Par ailleurs, il me semblerait judicieux d'attendre un retour d'expérience sur la forfaitisation de certains délits avant d'envisager

de l'auteur d'une infraction. Cette logique d'amende forfaitaire est en contradiction avec le principe d'individualisation de la peine, puisque chaque personne paye l'amende sans qu'il soit tenu compte de la situation. Enfin, le paiement d'une amende ne permet en aucun cas de mettre en place un mécanisme de prévention de la récidive à travers la compréhension de la portée de l'acte commis.

: La parole est à M. Jean-Luc Fichet. Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de la procédure de composition pénale. Aussi, le projet de loi prévoit de ne plus réserver le recours à cette procédure aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Une composition pénale pourrait ainsi être proposée pour tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue. En premier lieu, nous souhaitons rappeler que la composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme un mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves. La liste des infractions susceptibles d'être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999 par les lois de septembre 2002 et de mars 2004. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a encore étendu son champ d'application, désormais très vaste. Cette procédure peut en effet s'appliquer aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l'exclusion des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des délits d'homicide involontaire ou des délits politiques. En pratique, elle est surtout mise en oeuvre pour traiter des infractions simples en matière de délinquance urbaine de faible gravité, telles que les atteintes aux biens. Aussi, la préoccupation émise par notre commission, qui estime qu'« un grand nombre de petites infractions appelle une réponse pénale sans nécessairement mériter une audience devant le tribunal correctionnel », est déjà satisfaite dans les faits. En proposant la suppression de toute limite dans le seul objectif de faire du chiffre avec la réponse pénale, le projet de loi risque de dégrader ce dispositif. Le succès de la composition pénale ne dépend pas d'un effet de seuil, mais repose essentiellement sur la concertation entre le siège et le parquet. C'est la recherche d'un consensus minimum entre les magistrats du siège et du parquet sur les grandes lignes de conduite de la politique pénale locale qui favorise la réussite de la composition pénale.

n'a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction pénale, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ainsi que, le cas échéant, d'une ou plusieurs contraventions connexes. La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions, avec des sanctions adaptées, en application des dispositions de l'article 41-3 du code de procédure pénale. Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice causé, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer le dommage causé par l'infraction. Les dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale dix-huit mesures de composition pénale, parmi lesquelles figurent notamment le versement d'une amende, la réalisation de différents stages, l'interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement, la réalisation d'un travail non rémunéré ou encore l'injonction thérapeutique. Pour favoriser le recours à la composition pénale, le texte qui nous est soumis propose de supprimer la limitation aux délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus. La commission n'a pas jugé cette mesure inopportune

qui permettra au Parquet de recourir à la composition pénale pour tous les délits et non plus seulement pour ceux qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

Cela ne signifie pas que les faits les plus graves seront désormais punis d'une simple mesure de composition pénale, je tiens à le préciser. Il s'agit, par cette proposition, de donner davantage de souplesse

lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l'obligation de se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000euros. Une telle disposition est contradictoire avec la démarche de simplification et d'harmonisation qui inspire le projet de loi, en créant un nouveau seuil et une nouvelle procédure dérogatoire. Surtout, il est permis de considérer que la présente disposition s'écarte des exigences constitutionnelles. La phase de l'homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. À défaut, l'exigence d'un procès équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée. En matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle. L'exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l'action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d'un magistrat du siège, y compris sur des faits très graves. Il convient également de ne pas écarter l'hypothèse de la personne qui, après avoir donné son accord, n'exécute pas intégralement les mesures décidées dans le cadre de la composition pénale. Dans ce cas, la proposition initiale devient caduque. De telles mesures constituent des sanctions pénales. Leur exécution, même avec l'accord de la personne, requiert la décision d'une autorité de jugement.

avoir recours au juge du siège lorsqu'un accord a été trouvé entre la personne poursuivie et le procureur de la République ... Nous sommes effectivement dans un système dérogatoire.

issue du projet de loi comme étant contraire aux exigences constitutionnelles. Cependant, comme j'ai pu le dire au moment de la discussion générale, le projet de loi que je porte a été construit dans le respect des équilibres constitutionnels et procéduraux.

qui impose l'exigence de validation par le juge lorsque les mesures peuvent porter atteinte à la liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle le projet de loi limite la dispense de validation par le juge aux mesures qui peuvent être considérées comme ne portant pas atteinte à la liberté individuelle, à savoir l'amende de composition pénale, qui ne me semble pas porter atteinte à la liberté individuelle, et la remise de la chose ayant servi à commettre l'infraction ou en étant le produit. De plus, l'absence de validation par le juge ne concernera que les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, et à la condition que l'amende de composition ou la valeur de la chose dont le mis en cause devra se dessaisir n'excède pas

Le présent amendement vise donc à maintenir un assouplissement nécessaire et proportionné de la CRPC, très pratiquée et très appréciée des professionnels, en prévoyant un seuil intermédiaire de trois ans. Celui-ci paraît satisfaisant dès lors que la procédure de CRPC exige l'accord de la personne, l'assistance et la présence indispensable et obligatoire d'un avocat, ainsi qu'une homologation de la peine par un magistrat du siège. Bien évidemment, outre le seuil de trois ans demeure l'interdiction de prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue. Ainsi, pour vous donner un exemple, en cas de vol simple, qui est puni de trois ans d'emprisonnement, le maximum de la peine

impossibilité absolue » ou question touchant à l'ordre public. Or, dans la pratique, cette différence peut contribuer à un allongement considérable des débats, en particulier s'agissant de la constitution de la partie civile. Concrètement, il arrive que de vieux professeurs s'invitent à la barre pour commenter une affaire sans que le tribunal correctionnel puisse soulever l'exception préalablement. C'est pourquoi, afin de rationaliser les débats devant les tribunaux correctionnels, nous proposons cette nouvelle rédaction s'inspirant de celle qui est relative aux assises,

amendement tend à soulever une question technique relative au jugement des exceptions d'incompétence juridictionnelle et des exceptions d'irrecevabilité de constitution de partie civile. Ses dispositions se présentent comme une mesure de codification d'une jurisprudence de la Cour de cassation. Très sincèrement, la commission

selon lequel le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi d'incidents ou d'exceptions de procédures, doit joindre ces incidents à l'examen de fond de l'affaire, et doit statuer sur le tout dans une seule et même décision, sauf en cas d'impossibilité absolue ou lorsque la disposition contestée touche à l'ordre public. Concrètement, il me semble que ce texte satisfait l'exigence de bonne administration de la justice, en évitant que les différentes exceptions de nullité ne viennent paralyser la procédure pénale et ne soient en réalité utilisées à des fins dilatoires. Ainsi, le tribunal n'est pas obligé de renvoyer l'examen de l'affaire au fond dès lors qu'une nullité est soulevée, et il doit à l'inverse statuer sur le tout dans un même jugement. L'amendement que vous proposez vise à inverser ce principe pour les questions touchant à la recevabilité de partie civile et à la compétence du tribunal, en obligeant le tribunal en obligeant le tribunal à rendre un jugement sur ces exceptions avant d'examiner l'affaire au fond. Il me semble que cette complexification n'est pas justifiée. contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs de votre amendement, elle ne consacre pas la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en la matière. L'adoption de cet amendement obligerait le tribunal à statuer en deux étapes, ce qui me semble vraiment constituer une complexité procédurale supplémentaire, à laquelle je suis tout à fait opposée.

une solution probablement plus efficace serait de laisser le choix à la juridiction, lorsqu'elle pense que cela permet d'évacuer une vulnérabilité de la procédure et d'éviter des rebonds d'argumentation en cours d'audience ou des renvois, de se prononcer

décider de s'organiser comme il le souhaite. Il est déjà possible, au regard du droit existant, de les examiner avant le fond, ce qui est logique. C'est la raison pour laquelle je pense que votre observation, qui est tout à fait légitime, est déjà satisfaite en ce qui concerne

L'article 39 du projet de loi modifie le code de procédure pénale, notamment son article 388-5, qui prévoit la situation dans laquelle le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d'être assistés lors de leur audition par leur avocat. L'article 39 tend notamment à préciser le délai dans lequel l'avocat doit être convoqué et le délai avant l'accès au dossier. Le présent amendement vise à doubler les délais proposés par le projet de loi : de cinq à dix jours ouvrables pour ce qui concerne la convocation ; de quatre à huit jours ouvrables pour ce qui concerne l'accès au dossier. Il s'agit d'apporter de nouvelles garanties au principe du contradictoire, en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l'exercice des droits de la défense. Quel est l'avis de la

la commission ? La commission des lois est soucieuse d'assurer les droits de la défense, de préserver les intérêts de tous et de permettre aux avocats d'être présents dans les procédures.

Madame Deromedi, je partage totalement les observations de M. le corapporteur. J'ajouterai simplement que les délais proposés dans le texte constituent l'exacte reprise des règles aujourd'hui applicables en matière d'information judiciaire, qui prévoient les mêmes délais de quatre et cinq jours avant l'interrogatoire des parties par le juge d'instruction.

telle mesure figurait d'ailleurs dans le rapport remis par MM. Beaume et Natali à l'issue des chantiers de la justice. Comme eux-mêmes l'indiquaient, l'expérience des juridictions a montré que, très souvent, très souvent, certaines enquêtes, dans lesquelles les gardes à vue se terminent par un déferrement, sont ouvertes à l'instruction pour la simple et unique raison qu'une mesure de sûreté paraît opportune, alors que, en réalité il ne manque qu'un seul acte de pur complément à une enquête globalement achevée.

l'ouverture d'une information judiciaire va occuper du temps d'instruction sans bénéficier d'une quelconque plus-value de fond autre que celle d'attendre le versement de la pièce manquant au dossier. La procédure de comparution différée permettra ainsi, en l'attente du seul résultat de ces investigations, le prononcé d'une mesure de sûreté avant le jugement devant le tribunal saisi de l'action publique.

non pas à ouvrir une information judiciaire ou tout autre moyen pour compléter le dossier, mais à renvoyer immédiatement la personne devant le tribunal correctionnel, en lui fixant une date, plus ou moins lointaine- c'est un autre problème. Serait ainsi renvoyé devant le tribunal un dossier incomplet-

préciser devant vous que cette procédure de comparution différée est limitée dans le temps, ne pouvant excéder deux mois.

peut ne pas saisir un juge d'instruction. Il peut ne pas forcément demander une détention, surtout si celle-ci n'est motivée que sous la pression de l'opinion. Alors que nous devons promouvoir une autre politique pénale,

certes, éventuellement aller en détention provisoire, mais pas plus que deux mois. Dès lors que les pièces nécessaires pour le jugement seront réunies, elle passera en jugement. Par cette

présente une utilité, car le prévenu peut avoir intérêt à ce que sa situation soit examinée à l'occasion d'une audience unique. Une telle proposition, déjà approuvée au sein de l'institution judiciaire, est souvent pratiquée sous la forme d'une comparution volontaire du prévenu. Toutefois, en l'état du texte, les droits de la défense pourraient se trouver lésés, car le regroupement pourrait être imposé dans le cadre d'une procédure de comparution inadaptée aux circonstances en raison de critères d'urgence et de complexité différenciés. Par ailleurs, dans le cadre de la comparution sur procès-verbal, les dispositions relatives au délai d'information de dix jours de l'avocat et du prévenu sont inadéquates pour préparer une défense sur des dossiers multiples. Finalement, le regroupement des poursuites, présenté comme une avancée en termes d'efficacité et d'allègement des charges de la procédure et d'organisation des juridictions, pourrait constituer, dans certains cas, une atteinte aux droits de la défense.

sens souhaitable de conditionner le mécanisme du regroupement à l'accord du prévenu, afin d'assurer une conciliation plus satisfaisante entre l'efficacité recherchée des audiencements et les droits de la personne poursuivie.

si c'est utile à la procédure elle-même et si les dossiers sont liés. L'important est que le conseil du prévenu soit parfaitement informé et qu'il ait le temps de préparer la défense de celui qu'il assiste devant le tribunal correctionnel.

plusieurs affaires concernant un même prévenu et le citer à la même audience pour l'ensemble des faits pour lesquels il est poursuivi. En l'occurrence, il s'agit tout simplement de permettre au procureur, dix jours avant l'audience, de décider de regrouper des affaires pour lesquelles des citations n'auront peut-être pas encore été décernées ou renvoyées à des audiences ultérieures. Je ne suis pas sûr que, dans ce délai de dix jours, s'il y a plusieurs affaires différentes et parfois peut-être complexes, la défense ait le temps de préparer son argumentaire.